sur les entreprises de réseaux (IFER) mobile jusqu'en 2020 pour favoriser l'installation de nouvelles antennes de téléphonie mobile en zone de montagne, compte tenu des difficultés d'implantation propres à ces zones géographiques. Cette mesure a porté ses fruits, puisque, depuis le mois de juin 2017, selon les chiffres de la Fédération française des Télécoms, 5 114 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne, pour atteindre un total de 8 216 sites.

Je ne pense pas que la prorogation d'une exonération sur les antennes déjà existantes soit le meilleur moyen de promouvoir le déploiement de la couverture sur l'ensemble du territoire en réseau mobile, en particulier de la 4G. À ce jour, et c'est cela le plus important, les déploiements d'antennes dans les zones non couvertes sont d'ores et déjà exonérés au titre du mobile. les antennes installées dans les zones prioritaires qui sont, j'y insiste, bien identifiées, en lien avec les élus des territoires, bénéficient déjà d'une exonération d'IFER de cinq ans.

Il tend par ailleurs à rétablir une équité territoriale. Les différents systèmes d'exonération de certains sites dans les zones les plus rurales ou les plus montagneuses conduisent à une double peine et à une double « récompense Il vise enfin à insérer une approche environnementale de la taxation l'IFER. La multiplication des technologies déployées pose, avant la question fiscale, un problème environnemental. La 5G aura ceci de spécifique qu'elle sera énergiquement plus efficiente que d'autres technologies disponibles. Une fréquence donnée nécessitera, selon la technologie utilisée, plus ou moins d'énergie pour transporter le même volume de données. Aussi, il convient de voir comment inciter fiscalement les opérateurs à éteindre une technologie qui a un impact environnemental plus important qu'une autre.

? Si je partage le constat de Patrick Chaize sur la nécessité d'adapter l'imposition des principaux opérateurs en fonction de l'évolution de la couverture et de l'empreinte environnementale des technologies employées ou déployées, l'amendement me semble présenter une difficulté d'ordre technique. En effet, cet amendement vise à mettre en oeuvre un plafonnement de la taxe par décret, alors que le dispositif reste assez imprécis sur les conditions pouvant donner lieu à la minoration de la taxe, ainsi que sur l'ampleur de cette minoration. Ces éléments me conduisent à considérer que le dispositif

plus de lisibilité et de simplicité. Une concertation devrait être menée avec les acteurs au cours du premier trimestre de l'année 2021. Le Gouvernement émet un avis défavorable à ce stade, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas matière à améliorer le système de l'IFER, dont on sait la complexité et les défauts.

L'obtention de la note maximale conduirait le dispositif à bénéficier d'un crédit d'impôt, plus incitatif qu'une simple réduction d'impôt, dans la mesure où il peut faire l'objet d'un remboursement au contribuable si son montant dépasse le montant de l'imposition. Le montant de ce crédit d'impôt différerait selon le type de station installée. Ainsi, celles pour lesquelles un accord ou un avis de l'ANFR est requis, c'est-à-dire le dispositif de base, le crédit d'impôt correspondrait à 5 % du montant, tandis que, pour celles qui seraient uniquement soumises à déclaration, le crédit d'impôt serait intégral, le montant de l'IFER correspondant déjà à 10 % du montant pour pour un dispositif de base. De plus, le montant du crédit d'impôt pour les serait déterminé avant l'application des nombreuses réductions et exonérations, notamment pour l'installation dans les zones blanches, alors que celui pour les dispositifs de base serait calculé selon le montant définitif, si bien qu'il serait nul dans les cas où les stations bénéficient d'une exonération. Par conséquent, dans les zones à exonération, notamment les zones blanches, les opérateurs seraient incités à installer des plutôt que des BTS (). Enfin, comme il est d'usage pour les crédits d'impôt d'initiative parlementaire, il convient d'ajouter un paragraphe III à l'article additionnel, prévoyant que ce crédit d'impôt ne s'applique qu'en déduction des sommes, c'est-à-dire

demande le retrait

correspondant aux employés concernés par le télétravail. Mme Lavarde a justement expliqué cet après-midi que les entreprises étaient les principaux acteurs du financement du système

Plus fondamentalement, enfin, le versement mobilité doit être appréhendé non pas comme une redevance, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire un impôt assis sur la masse salariale, qui permet de contribuer au financement des transports publics.

cet amendement. Le versement mobilité est dû par les entreprises, dès lors que la collectivité compétente le décide, et il ne varie pas en fonction de la part des salariés qui ont recours aux transports collectifs. Il n'est pas même conditionné par la desserte de l'entreprise par

à qui on a demandé de mettre leurs salariés en télétravail ont dû, dès lors qu'elles ont signé des accords, déployer des ressources matérielles

Le transport en Île-de-France est totalement régi par l'État, avec des poupées russes de sociétés d'État qui s'endettent sans tenir compte ni des collectivités locales ni, surtout,

qui avait pour objet de fixer les principes généraux de la fiscalité du centre de stockage industriel en couches géologiques profondes des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue

progressé sur le système de fiscalité que supportera Cigéo. Nous sommes d'accord avec le Gouvernement sur les conclusions et les principes généraux édictés par les trois inspections qui ont travaillé sur ce sujet et qui sont à l'origine de l'amendement qu'il a présenté,

Il est donc nécessaire d'en tenir compte dans la taxe de stockage que les producteurs de déchets nucléaires doivent acquitter en contrepartie de cet effort que deux départements, la Haute-Marne et la Meuse, ont consenti en acceptant ces déchets. Le second point de désaccord est moins important. Nous considérons que la répartition de cette taxe entre les collectivités locales de proximité, le département, la région et accessoirement l'État doit être fixée par la loi pour que le débat soit transparent. Nous avons donc déposé cet amendement,

bien montré qu'il y avait une complexité, elles n'ont pas tranché. Si l'on veut que le dispositif avance, on a besoin aujourd'hui que le Parlement soit éclairé pour voter, sur la base de cet amendement, en connaissance de cause.

Cet amendement ne ferme aucune porte. Il vise à renvoyer un coefficient à un décret en Conseil d'État, qui peut être négocié, et la répartition entre les collectivités à la loi. Il a l'immense mérite d'obliger le Gouvernement à prendre ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle je demande à mes collègues

et d'entamer un vrai débat avec les populations et les élus. Cette affaire n'a que trop duré. Je ne sais pas comment elle sera tranchée ; en tout état de cause, nous avons toutes et tous intérêt à engager un débat démocratique sur ce sujet. La parole est à M. Bruno Retailleau,

qui s'appliquerait de manière uniforme, quelle que soit la durée de détention du bien, à l'exception des deux premières années. Pour les plus-values à très court terme, un taux supérieur serait conservé. Cette mesure simplifierait opportunément le régime d'imposition en vigueur et renforcerait son efficacité. Ce serait une bonne

Ses conclusions, rendues en 2015, citaient le régime d'imposition des plus-values de cessions immobilières parmi les exemples de fiscalité particulièrement complexe et peu lisible. Il me faut aussi convenir que supprimer tout abattement pour durée de détention est une idée intéressante et séduisante.

écologique. Le nombre de ces logements vacants paraît injuste et absurde au regard des besoins. D'après la Fondation Abbé Pierre et le Secours populaire, la crise sanitaire a exacerbé les besoins 8 millions de personnes sont en situation de mal-logement en France et 900 000 personnes ne disposent pas d'un logement individuel. Le Secours populaire a vu le nombre de personnes qu'il aide augmenter de 45 %. Cet amendement vise donc à exprimer l'ambition annoncée au mois de février dernier par le ministre chargé de la ville et du logement : inciter les propriétaires de logements vides en zone tendue à les louer.

une vision aussi uniforme, pour ne pas dire dogmatique, des raisons pour lesquelles un certain nombre de biens ne trouvent pas preneurs ou restent vacants. On a mille et une situations

un désintérêt pour les opérations de réaménagement de parcelles bâties, un abandon des politiques publiques en matière d'accession à la propriété et de location, et des contrôles fiscaux en chaîne. Alors que le Gouvernement a lancé des opérations de recyclage urbain dans le cadre des programmes Action coeur de ville et Petites villes de demain, et que les finances des collectivités sont lourdement touchées par la crise, la lecture imposée par l'administration fiscale ne paraît ni opportune ni juste. Cet amendement vise donc à clarifier et à affermir l'application de la TVA sur marge dans le cadre des opérations de viabilisation des terrains à bâtir, dans le respect du droit européen.

en déduisant de la valeur réelle des biens et droits immobiliers le montant de la totalité des dettes contractées par la société à prépondérance immobilière. Dans un souci d'équité fiscale et de limitation des abus, nous proposons de mettre fin à la possibilité de déduire les montants des emprunts et des comptes courants de la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus.

qui réduit les recettes de l'État et des collectivités locales. S'agissant de ces dernières, on peut penser qu'en supprimant cette possibilité d'optimisation un certain nombre de transactions immobilières

Cet amendement a pour objet d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens ayant acquis les locaux dans lesquels ils assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours. Il s'agit ainsi de mettre fin à une rupture d'égalité entre deux types de structures ayant le même objet : les professionnels libéraux exerçant dans des structures appartenant aux collectivités locales bénéficient de conditions d'exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées, qui sont par ailleurs soumises aux mêmes obligations d'accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires. J'ai présenté un amendement similaire l'année dernière. En cette période où

pour la rénovation urbaine (ANRU), la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d'exonération de taxe foncière si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50 % de logements sociaux. Cette règle a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2017, sur proposition de certains élus locaux qui, s'inquiétant des pertes de recettes fiscales liées à ces exonérations, souhaitaient limiter la concentration des logements sociaux sur leur territoire, sachant que ces logements étaient déjà nombreux. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles et qu'il convient que les efforts de construction et de mixité soient bien partagés, il existe des situations où la reconstruction sur place s'impose, en raison de spécificités particulières. Cet amendement vise ainsi à permettre aux élus locaux de déroger à la règle, s'ils le souhaitent. La

taxe foncière. Il s'agit de proposer une exonération de taxe foncière pour les constructions sur des bâtiments démolis qui en avaient déjà bénéficié,

font l'objet d'une compensation par l'État, laquelle se trouve justifiée en raison de leur caractère obligatoire. Or l'article 1 384 G fait référence aux exonérations des articles 1 384 et suivants.

Cet amendement vise à répondre à un problème matériel lié au calendrier électoral. En effet, la prorogation d'une convention d'utilisation de la TFPB, permettant un abattement de 3 % pour les logements locatifs sociaux de la politique de la ville, doit intervenir avant le 1 octobre de l'année au cours de laquelle la convention arrive à échéance pour permettre le maintien de l'abattement pour l'année suivante. suivante. Nous proposons, par dérogation aux règles de délai prévues par la loi, de décaler au 30 juin 2021 la date limite de signature de la convention pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de

Cet amendement vise à corriger une injustice et à faciliter le financement d'infrastructures de transport, qui est très délimité. Lorsqu'une gare

les taxes existantes- taxe communale additionnelle aux droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière et autres taxes communales -dans un périmètre restreint autour de ces infrastructures, afin de mieux financer ces investissements particulièrement dispendieux.

d'une infrastructure de transport collectif. Si l'on peut comprendre qu'une partie de la plus-value créée par le développement d'infrastructures de transports revienne à la collectivité,

faciliter la requalification du tissu existant et d'attirer une nouvelle population. Afin de favoriser des opérations d'accession à la propriété dans ce cadre, il est proposé que les conseils départementaux, s'ils le souhaitent, puissent intervenir en soutien des villes concernées, en exonérant de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière les ventes de logements, sous réserve du respect des conditions qui s'imposent aux organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) en matière d'accession sociale à la propriété, qu'il s'agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement.

libérant ainsi les acquéreurs accédant à la propriété du foncier. Ces opérations, encadrées par un mécanisme anti-spéculatif strict, se développent sur l'ensemble du territoire, avec l'appui d'un certain nombre de collectivités locales volontaires.

tour ses droits à un ménage. Chacune de ces mutations est en principe soumise à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement. La loi de finances rectificative pour 2016 a en partie remédié à ce cumul de taxes, en prévoyant, dans certaines situations, une exonération des droits sur la deuxième mutation. Cela ne semble toutefois pas suffisant. Afin d'encourager ce type d'opération,

est devenu un outil pour les collectivités voulant agir au service de l'accession à la propriété des ménages à revenus très modestes. Il a vocation à se développer dans tous les territoires, dès lors qu'il y a un enjeu de maîtrise du foncier.

Cela freine à la fois la réhabilitation des logements anciens, souvent situés en centre-ville ou centre-bourg et incite à la construction de logements nouveaux, participant ainsi à l'artificialisation des sols. Cet amendement vise donc à permettre aux conseils départementaux d'instituer un abattement sur l'assiette de la taxe de publicité ou de droit d'enregistrement, au cas où les travaux réalisés dans un logement ancien dépassent 25 % de la valeur du logement pour lequel l'acquéreur s'engage à réaliser les travaux en question.

Cet amendement vise à ce qu'un conseil départemental puisse- c'est bien une faculté, monsieur le rapporteur général, et non une obligation -réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement jusqu'à 0,7 %, en cas de mutation d'un immeuble bâti lorsque l'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à réaliser les travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production et à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257. Il s'agit là d'une recommandation figurant au rapport «

Face aux difficultés d'accès au logement des personnes les plus démunies, l'Union sociale pour l'habitat a proposé un dispositif visant à développer, avec le concours d'associations agréées d'intermédiation locative volontaires, l'intervention des organismes d'HLM dans le parc privé, afin de libérer des places d'hébergement. En effet, si des efforts sont faits chaque année pour multiplier ces places, ils ne sont cependant jamais à la hauteur des besoins. L'intervention du secteur HLM est donc à encourager.

Selon les chiffres de la ministre déléguée chargée du logement, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et par personne, contre 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit d'hôtel.

Pour soutenir ce dispositif, il est proposé une exonération facultative, sur décision des conseils départementaux, au profit des acquisitions de logements réalisées, dans ce cadre, par les organismes d'HLM. L'exonération serait subordonnée à l'engagement de l'organisme de louer ces logements à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative pour une durée d'au moins six ans. Le non-respect de cet engagement sera bien sûr sanctionné.

situés outre-mer. Cette cotisation est assise sur les loyers encaissés au cours de l'année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité. Le taux maximal applicable est de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.

serait d'autant plus justifiée que les barèmes de plafonds de ressources applicables dans les départements concernés conduisent à majorer le montant global de ce supplément par rapport à la France hexagonale.

redevances et produits du supplément de loyer de solidarité qu'ils perçoivent au titre de leurs logements à usage locatif et de leurs logements foyers. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, les organismes de logement social bénéficient déjà d'un plafonnement du taux de cotisation principale

à certaines obligations de paiement, notamment l'obligation de payer des acomptes au fur et à mesure de la réalisation des prestations, à l'interdiction des paiements différés et à la distinction entre la rémunération des prestations d'exploitation et de maintenance et le paiement de la construction. Certes,

absolument stratégique de l'articulation entre les établissements de santé privés et les hôpitaux publics. Or ces deux

exclut les sites d'enfouissement des déchets dangereux du bénéfice d'une mesure qui leur est applicable d'après la loi de finances pour 2020. L'exonération ne peut intervenir qu'après la parution d'un arrêté préfectoral, dont chacun sait qu'elle peut prendre plusieurs années.

exonération. Il faut être clair et ne pas chercher à offrir en catimini, par l'adoption d'un amendement, un allégement de fiscalité locale aux entreprises de stockage de déchets dangereux, qui ne serait ni négocié ni compensé.

dans les deux types d'installations. De plus, un site peut être qualifié de multifilières et comprendre une zone destinée au traitement et au stockage des déchets dangereux et une autre destinée au traitement et au stockage des déchets non dangereux. l'article 42 présente des difficultés qui feront obstacle à son application. Cet amendement vise à y remédier et à rendre le dispositif compatible avec le principe de l'unité d'évaluation foncière. Son adoption garantirait que le changement de méthode bénéficiera à tous les terrains, bâtiments et installations foncières concourant à l'activité de stockage des déchets.

raisons. Pendant plusieurs années, les collectivités territoriales pouvaient décider d'une exonération de taxe foncière en faveur de certains sites de stockage de déchets non dangereux. pour 2020, le rapporteur général de l'Assemblée nationale, M. Giraud, a fait adopter un amendement visant à transformer cette exonération en nouvelle modalité de calcul de la valeur locative des sites.

Ce soir, il est proposé au Sénat d'étendre cet allégement de fiscalité au stockage des déchets dangereux.

Cette exploitation en différents casiers est prévue dans la réglementation. La période d'exploitation commerciale d'un casier commence à la date de réception des premiers déchets et se termine à la date de réception des derniers déchets dans celui-ci. La fermeture du casier équivaut donc à la fin de son exploitation commerciale. En revanche, la délivrance d'un arrêté préfectoral de post-exploitation est sans lien direct avec l'exploitation commerciale du site : c'est une procédure administrative, qui peut prendre plusieurs années en fonction des délais liés à la prise à la prise de l'acte administratif. La fermeture du casier correspond donc à la période pendant laquelle l'exploitant ne peut plus en tirer aucun revenu.

conformément aux dispositions de l'article 1522 du code général des impôts, le montant total de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dû par le contribuable est établi d'après le revenu cadastral net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. S'agissant d'une taxe, ces sommes ne rémunèrent pas une prestation, mais financent un service public, sans corrélation avec la quantité de déchets produits par les foyers. Or si une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, avec l'unique possibilité pour la collectivité ou l'EPCI de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM. Cette possibilité indifférenciée ne répond pas à la problématique spécifique des ménages modestes. En outre, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s'appliquent pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ailleurs, dans les cas où le propriétaire récupère la TEOM auprès de son locataire, ce dernier ne peut, en tout état de cause, que bénéficier des dégrèvements prévus pour son propriétaire, ce qui ne correspond pas à sa situation personnelle. la mise en place d'une part incitative de la TEOM en application de l'article 1522 du code général des impôts peut amoindrir l'effet pénalisant pour les ménages modestes, elle ne elle ne permet pas d'intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d'habitation. dans un souci de justice sociale et de respect de l'autonomie fiscale, cet amendement vise à donner la faculté aux collectivités locales et à leurs groupements de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, et les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes.

Rambaud vise à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui seront bénéficiaires des 750 millions d'euros de crédits ouverts par la quatrième loi de finances rectificative sous la forme d'avances remboursables dont les conditions d'application seront précisées par décret, d'inscrire ces avances en recettes de leur compte administratif pour 2020. Dans la mesure où cette avance remboursable répond à des pertes de recettes fiscales et tarifaires que subissent les AOM en 2020, il est logique de les autoriser à rattacher le montant de l'avance à l'exercice 2020. Quel est l'avis de la

Cette modification n'affecterait pas les industriels, mais elle permettrait de modifier la répartition pour nos communes. Depuis 1910,

Ce dispositif temporaire s'appliquerait aux déclarations effectuées au titre des années 2021 et 2022. Il s'inscrit dans la stratégie que le Gouvernement a présentée le mois dernier pour accélérer la sortie du glyphosate des pratiques agricoles d'ici à 2022,

le crédit d'impôt proposé est limité par la notion d'activité « principale » qui risque d'exclure de nombreux exploitants agricoles qui s'engageraient à ne pas utiliser de glyphosate. En matière fiscale, et sans précision complémentaire, l'activité principale se définit généralement comme l'activité générant la part prépondérante de chiffre d'affaires au sein de l'exploitation. En outre, l'amendement actuel n'introduit aucune notion de proportionnalité : soit l'activité principale de l'exploitation est éligible et l'entreprise perçoit un crédit d'impôt pouvant